Cette somme très importante doit nous faire prendre conscience de l’ampleur des dégâts matériels, économiques et sociaux. Pour les seules infrastructures publiques, il faudrait 1 milliard d’euros. Cet amendement vise à appeler à la mise en œuvre d’un plan de reconstruction ambitieux dès l’année 2025, à hauteur de 2,1 milliards d’euros. Cette année 2025 sera cruciale pour la reconstruction de la Kanaky Nouvelle Calédonie. Agissons dès maintenant ! L’amendement n° I 752 est un amendement de repli. Il tend à une contribution à hauteur de 850 millions d’euros pour l’année 2025. Quel

Depuis près de deux ans, les travailleurs du social et du médico social se mobilisent pour l’élargissement de la prime Ségur. Après d’âpres négociations, le 4 juin 2024, la CGT, la CFDT, Force ouvrière et SUD ont signé l’accord avec les confédérations d’employeurs permettant,

entre 92 400 et 215 000 professionnels de secteurs médico social et social du privé non lucratif avaient été exclus du Ségur. Cette mesure de justice est donc une bonne nouvelle, à la condition que l’État compense aux départements l’intégralité du surcoût occasionné. L’État ne peut engager les départements chefs de file sur la compétence du médico social et se désengager ensuite lorsqu’il s’agit de compenser financièrement l’extension de la prime Ségur. Notre amendement vise à mettre l’État devant ses responsabilités, en refusant le transfert de 170 millions d’euros sur les départements.

Canalès. Il vise à renforcer les moyens dédiés au contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant par les services départementaux de protection maternelle et infantile. Aujourd’hui, selon des données de l’inspection générale des à ce contrôle dans toute la France. Afin de renforcer le contrôle de la qualité de l’accueil dans les établissements d’accueil du jeune enfant, cet amendement tend à un prélèvement sur recettes de l’État pour porter à 150 ETP le nombre de postes dédiés dans notre pays. Quel

à 150 millions d’euros, ce qui permettra tout de même aux organismes de l’audiovisuel public de disposer d’un niveau de financement supérieur à celui de 2023. Au regard des moyens nouveaux qui ont été mobilisés en 2024 et de la situation budgétaire, il nous est apparu que cet effort était à la mesure des capacités de l’audiovisuel public et de France Télévisions.

Je me fais ici la porte parole du président de la commission de la culture, du rapporteur spécial et du rapporteur pour avis des crédits de l’audiovisuel, qui sont beaucoup plus compétents que moi pour pour parler de ces sujets. Mes trois collègues estiment qu’il est possible de porter l’effort demandé aux sociétés de l’audiovisuel public à 15 millions d’euros de plus que l’effort initialement

La mesure aurait un rendement estimé à 4 milliards d’euros par an et permettrait à l’ensemble des foyers déclarant un revenu inférieur à 55 200 euros de payer une contribution moins élevée que lorsque celle ci était forfaitaire. Je ne sais

un pouvoir démocratique.

mettre en place une contribution affectée beaucoup plus progressive et, surtout, fonction du niveau de revenus des citoyens, dont le montant et l’affectation seraient contrôlés par un organisme indépendant, sur le modèle allemand.

aussi un message politique : celui d’une lassitude à l’égard de l’omniprésence de la publicité et de l’incitation à la consommation. Nous ne pouvons accepter y soient consacrés, alors que, dans le même temps, on a demandé à France Télévisions d’appliquer, depuis quatre ans, un plan d’économies de 190 millions d’euros. Allons chercher les moyens là où ils se trouvent ! La publicité peut être une bonne

son rôle est très limité, car son conseil d’administration ne fait qu’avaliser des décisions déjà prises, soit par le Gouvernement, soit par l’administration, au point que la question du financement des infrastructures de transport

à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en 2025, par rapport au niveau qui figurait en loi de finances initiale pour 2024. Le financement des infrastructures de transport répondant à une logique de temps long, il est en effet nécessaire d’éviter une baisse trop brutale des moyens

Cet affaiblissement s’explique principalement par une chute d’un ordre de grandeur de 700 millions d’euros du montant de TICPE affecté à l’agence pour 2025. Or cette recette est assise en grande partie sur le secteur des transports. Cette désaffectation constitue donc une fuite des impôts payés par ce secteur vers le budget général de l’État. Ce mouvement est contradictoire avec la nécessité de renforcer le report modal et d’assurer la décarbonation des mobilités. La trajectoire de financement de l’Afit France pour 2025 s’inscrit en effet, pour l’instant, dans le scénario de cadrage budgétaire du Conseil d’orientation des infrastructures (COI), et non dans son scénario de planification écologique, qui est pourtant la feuille de route sur ce sujet.

Et la France ne s’en portera pas plus mal

pour financer le douzième programme des agences de l’eau et accompagner les collectivités locales, déjà sous très forte contrainte budgétaire, afin qu’elles ne supportent pas seules la charge financière des projets liés à la gestion de l’eau sur le territoire. En outre, le plafond mordant

Si les ressources sont supérieures aux dépenses attendues, alors nous devrions nous réjouir et réfléchir à la façon dont les agences de l’eau peuvent développer leurs actions, par exemple en aidant les acteurs responsables de la pollution de l’eau à transformer leurs pratiques, ou bien, à l’inverse, baisser le coût de l’eau pour les particuliers

I 1999, présenté par Mme de Marco,

Le déplafonnement de la taxe versée à l’Association pour le soutien du théâtre privé serait donc contraire à cette disposition de la LPFP. Et elle ne serait justifiée par aucune circonstance spécifique. J’émets donc

proposons que le tarif unitaire de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, déterminé en fonction de la puissance administrative du moteur du navire, s’applique dès le premier cheval à partir d’une puissance administrative de 26 chevaux, soit un moteur essence de 250 chevaux, au lieu de 100 chevaux comme il est actuellement L’abattement sur les cinq premiers chevaux ne s’applique plus qu’aux petits moteurs entre 6 chevaux et 25 chevaux. De plus, l’amendement tend à augmenter de 50 % les tarifs unitaires à partir de 26 chevaux. Ce faisant, il est ici proposé de renforcer le caractère environnemental de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel.

examinés, nous proposons de déplafonner la taxe sur la billetterie affectée au Centre national de la musique (CNM), dont le plafond est aujourd’hui fixé à 50 millions d’euros. Le CNM, qui a été créé en 2020, a pour vocation d’être le centre de toutes les musiques et de garantir la diversité,

Cette taxe constitue la principale source de financement du CNM. Ses recettes sont amenées à croître dans les prochaines années, comme l’indique le contrat pluriannuel d’objectifs et de performance

vise à préciser le rendement prévisionnel pour 2025 de la contribution annuelle à la charge des professionnels de santé affectée à la

paris sportifs en ligne de la Française des jeux affecté amendements visaient à déplafonner intégralement les taxes affectées à l’Agence nationale du sport. L’objectif est de rétablir une redistribution équitable des ressources pour soutenir durablement les politiques sportives,

Cet amendement vise à augmenter de 40 millions d’euros le plafond de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie, afin de respecter la trajectoire pluriannuelle définie lors du projet de loi de finances pour 2024, qui prévoyait le maintien de la TCCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027. En échange, il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros annuels sur le fonds de roulement.

Bien que nous soyons conscients de la nécessité de redresser les comptes publics, il est crucial de préserver les moyens d’action des CCI, qui jouent un rôle majeur dans le développement de notre tissu économique, tant local que national. Les

l’avis du Gouvernement ? J’émets un avis favorable sur l’ensemble de ces amendements. On me dit qu’il y a une différence rédactionnelle entre ce bloc d’amendement et les suivants…

et le Gouvernement. Il se justifie par une volonté de lissage des 53 millions d’euros de baisse restants sur les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait dû afficher une baisse de 13,25 millions d’euros, et non de 20 millions d’euros. Pour donner de la visibilité budgétaire

Je vous remercie

La trésorerie du CNC constitue la contrepartie d’engagements inhérents à son activité, ainsi que de risques avérés, notamment sur le plan contentieux. En effet, le CNC verse environ 750 millions d’euros d’aides chaque année à l’ensemble de la filière du cinéma et de l’audiovisuel. Ainsi, la trésorerie permet d’assurer que le Centre peut effectivement verser les aides attribuées, lorsque ses bénéficiaires en font la demande. Dans ce contexte,

D’ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport de 2023, l’inspection générale des finances, dans sa revue de dépenses de 2024, et les services de Bercy eux mêmes ont tous partagé ce constat objectif : le montant de 450 millions d’euros est le seuil maximal.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Dans ce rapport, les inspections recommandent d’engager un travail de rationalisation des exonérations d’assiette de la taxe d’apprentissage, en particulier celles qui visent certains employeurs en raison de leur statut juridique.

locales. Depuis 2019, les agences de l’eau sont déjà soumises à un plafond annuel légal de redevance, dit plafond mordant. Ce mécanisme est d’ailleurs questionné dans un rapport sénatorial qui indique qu’il est vécu comme une captation illégitime des ressources affectées à l’eau au profit du budget de l’État. Dans un souci de compromis, ce sous amendement vise à réduire de moitié le prélèvement envisagé, en le portant à 65 millions d’euros, au lieu des 130 millions d’euros initialement prévus par le Gouvernement.

En ciblant spécifiquement les décollages de nuit, particulièrement nuisibles au sommeil et à la santé des riverains, cet amendement tend à inciter les compagnies aériennes, notamment, à limiter ces vols. En modulant la taxe selon l’horaire, nous donnons un signal économique fort aux aérodromes pour qu’ils réduisent l’impact nocturne des nuisances sonores. De plus, cette mesure permettrait d’augmenter la prise en charge des travaux d’isolation phonique à 100 %. favoriserait l’accès à l’insonorisation pour les ménages les plus modestes et permettrait d’élargir progressivement le périmètre des logements éligibles.

fait l’objet depuis sa création de nombreuses critiques. À l’origine fixée à un montant de 90 euros, la contribution est indexée sur l’inflation et atteint 103 euros en cette rentrée 2024, soit un niveau inédit. Collectée par les Crous et redistribuée partiellement aux universités, la CVEC est payée chaque année par les étudiants. Et c’est bien ce mode de fonctionnement que nous ne partageons pas : alors que la précarité étudiante ne cesse de s’accroître et que les files aux distributions alimentaires ne se sont jamais arrêtées, les étudiants ne devraient pas avoir à payer pour le fonctionnement de nos universités.

devrait atteindre 176 millions d’euros en 2025 en faveur des établissements d’enseignement supérieur et à destination du réseau des œuvres universitaires et scolaires. Or

– bac pro, BTS, master, etc. –, afin d’éviter une déperdition de sens de ce dispositif. D’autre part, il a pour objet de redynamiser la contribution supplémentaire sur l’apprentissage, pour prendre en compte la hausse du développement de l’apprentissage depuis 2014. On le sait, et

pour les employeurs ayant conclu un contrat d’apprentissage avec un apprenti relevant d’un établissement d’enseignement supérieur de droit privé à but lucratif. Mes chers collègues, je souhaite vous alerter sur ce sujet bien précis des établissements privés à but lucratif. En effet, un rapport de la mission d’information sur l’enseignement supérieur privé à but lucratif déposé en avril dernier à l’Assemblée nationale souligne les dérives et le manque de régulation à la suite de l’essor de ces établissements. Cet essor s’explique en grande partie par le recours massif aux aides à l’apprentissage, qui, selon la Cour des comptes, ont globalement coûté 16,8 milliards d’euros à l’État. Le privé lucratif a entraîné de trop nombreuses familles dans des situations extrêmement difficiles. Nous devons légiférer pour limiter les effets d’aubaine dont tirent profit ces établissements. Monsieur le ministre, vous l’avez dit vous même lors d’une audition au Sénat, vous êtes prêt à agir pour réguler l’enseignement privé lucratif. Aussi, régulons ! Je pense que nous pouvons mener un travail transpartisan sur ce sujet,

la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) diminue de 300 millions d’euros en 2025, même si Action Logement, de son côté, n’y contribuera plus. Nous sommes dans une situation où les bailleurs sociaux sont de plus en plus affaiblis et où leurs finances dépendent en très grande partie des loyers de leurs locataires.

réduction de loyer de solidarité (RLS) serait un signal positif de confiance pour le secteur. Malheureusement, c’est tout l’inverse. Monsieur le ministre, les bailleurs sociaux sont en colère,

l’État s’est engagé à mettre en place un cadre de financement favorable à la production de logements sociaux. Cela s’est traduit par un montant de contribution des bailleurs sociaux à la CGLLS de 75 millions d’euros. Pour rappel,

M. le ministre. Il s’agit de l’extension du mécanisme d’avances remboursables de court terme aux collectivités d’outre mer non couvertes actuellement en cas de difficultés de trésorerie.

Depuis sa création en 2012, l’enveloppe du CAS Facé n’a jamais été revalorisée, restant figée à 360 millions d’euros. Dans un contexte où les territoires ruraux font face à des défis croissants, notamment liés à l’augmentation des aléas climatiques et à la transition énergétique, cette stagnation budgétaire aggrave une fracture territoriale déjà profonde. Le rôle du CAS Facé est crucial. En remplaçant la contribution des gestionnaires de réseaux de distribution par une fraction de l’accise sur l’électricité uniformisée à l’échelle nationale, cette réforme met fin à la logique de péréquation qui soutenait jusqu’à présent les zones les plus vulnérables. Comment justifier une telle mesure, alors que les territoires doivent renforcer leurs infrastructures face au défi climatique et énergétique ? Cette réforme non seulement fragiliserait la pérennité des aides à l’électrification rurale, mais pourrait conduire à la suppression pure et simple du CAS Facé. L’absorption de ses crédits dans le budget général de l’État serait une perte considérable pour nos Pour finir, c’est un recul pour les réseaux de distribution ruraux, puisque la réforme aboutirait à une décorrélation entre les aides allouées et les besoins réels des territoires. Alors que les réseaux publics d’électricité en zone rurale doivent faire face à des investissements massifs pour répondre à la montée en puissance des déchets d’énergies renouvelables et des usages électriques, cette réforme les prive de garanties de financement adaptées à leurs spécificités. En outre, elle rompt le lien avec le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe), qui finance jusqu’à présent de manière cohérente les réseaux publics, qu’ils soient urbains ou ruraux. Cette rupture pourrait entraîner des risques juridiques importants, fragilisant davantage les zones rurales. Ne nous y trompons pas, cette réforme n’est ni une simplification ni une solution pérenne. Elle constitue une menace directe sur nos

l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité

Cet amendement vise à supprimer l’article portant sur les relations financières entre l’État et la sécurité sociale, qui comprend, d’une part, la neutralisation des décisions en matière de politique de l’emploi sur les comptes de la sécurité sociale et, d’autre part, la ponction de l’État sur les comptes de l’Unédic, pour financer son désendettement désordonné.

des allégements généraux pour un rendement brut de 5,1 milliards d’euros en moins. Parce qu’elle entraîne mécaniquement une hausse du montant des cotisations patronales acquittées et une réduction des bénéfices des entreprises, cette mesure a pour conséquence d’amoindrir le rendement de l’impôt sur les sociétés,

Le Gouvernement a fait le choix de maintenir en 2025 l’affectation du rendement net de la réforme des allégements généraux à la sécurité sociale, en neutralisant cependant ses effets sur les recettes au budget général. pour 2025, issu des travaux de la commission mixte paritaire, prévoit désormais un rendement brut de 2 milliards d’euros et un rendement net de 1,6 milliard d’euros au titre de la réforme des allégements généraux,

ce seront 3,35 milliards d’euros qui seront prélevés pour financer la création de France Travail. Cette ponction, qui pourrait atteindre un montant compris entre 3,5 milliards d’euros et 4 milliards d’euros en 2026, selon la lettre de cadrage envoyée par le Gouvernement aux partenaires sociaux,

Je profite de l’examen de ces amendements sur l’Unédic pour rappeler que le Gouvernement fait des choix budgétaires qui ne sont pas neutres. Je pense en particulier à la question de l’indemnisation des travailleurs transfrontaliers. En 2023, quelque 77 000 allocataires étaient indemnisés par l’assurance chômage en France, alors qu’ils avaient travaillé et cotisé dans un pays frontalier. Sur les quelque 2,5 millions de chômeurs indemnisés, c’est peu, mais c’est 50 % de plus par rapport à 2020. En principe en principe seulement ! –, un système de compensation financière par les États dans lesquels les travailleurs ont cotisé est prévu par la réglementation européenne. Toutefois, selon les gestionnaires du régime, les dépenses à la charge de l’Unédic sont nettement supérieures aux remboursements. En 2023,

La logique voudrait que le Gouvernement se mobilise pour récupérer 800 millions d’euros d’indus auprès d’autres États membres de l’Union européenne. Les négociations

n° I 589. Les missions régaliennes de sûreté sécurité dans les aéroports français sont réalisées par les exploitants d’aéroport. Ceux ci reçoivent en contrepartie des recettes fiscales destinées à couvrir le coût de ces missions : le tarif de sûreté sécurité (T2S). Pendant la crise sanitaire, les recettes de T2S ont fortement diminué, tandis que les dépenses de sûreté sécurité sont restées stables. Par conséquent, l’État a consenti aux aéroports des avances, pour un total de 700 millions d’euros. Afin de favoriser un remboursement de ces avances sans pour autant augmenter trop fortement le montant du T2S, qui serait répercuté sur le prix du billet, l’article 39 prévoit d’augmenter le ticket modérateur du T2S. Compte tenu de ce contexte, cet amendement vise à revenir pour moitié sur cette hausse du ticket modérateur du T2S, en le limitant à 8 % du montant des dépenses de sûreté sécurité. L’amendement

Cet amendement vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à abandonner tout ou partie des créances détenues par l’État sur la compagnie aérienne Corsair, pour un montant de 80 millions d’euros en capital.

la loi de finances pour 2024 et la loi du 9 avril 2024 visant